Monsieur le président,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

Monsieur le ministre, mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est une voix du Sénat écoutée, tolérante qui s'est éteinte avec François Fortassin. C'est une figure charismatique et chaleureuse de la Bigorre qui s'en est allée.

une maladie qui l'avait affaibli, mais ne l'empêchait pas d'être toujours présent au Sénat, de participer aux travaux de notre bureau, avec la simplicité, l'accessibilité et la chaleur qui ont toujours Cet amoureux de la vie, de son pays et de son territoire nous manque. Oui, c'est avec émotion que nous avons appris sa disparition le 15 mai dernier, au lendemain même de la cérémonie d'installation du Président de la République, dont il avait parrainé la candidature et qu'il avait soutenu,

à l'occasion d'une émouvante cérémonie au coeur de sa commune natale de Sarp au milieu de ses proches et de ceux qui lui étaient chers. J'étais accompagné J'étais accompagné de plusieurs membres du bureau du Sénat, dont François Fortassin était membre depuis 2008, nos collègues Françoise Cartron

Cet hommage trouve aujourd'hui, après la reprise de nos travaux en séance publique, son prolongement dans notre hémicycle. François Fortassin représentait le département des Hautes-Pyrénées au sein de notre assemblée depuis depuis le 3 mars 2001, date du décès de François Abadie, dont il était le suppléant depuis 1983. Nous étions alors à quelques semaines des élections sénatoriales. François Fortassin était un humaniste. Ses convictions républicaines et laïques trouvaient leur expression dans les valeurs du radicalisme, qu'il portait haut et fort, avec un mélange de douceur, de sens de l'écoute, mais aussi de force. Il sera toujours fidèle à ces valeurs, qu'il retrouva au Sénat au sein du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, et sur la scène politique parmi les radicaux de gauche. C'est, disait-il, « le parti le parti qui correspond le mieux à ma sensibilité : on y privilégie l'humanisme et l'épanouissement individuel. J'ai été influencé, lors de mes études d'histoire, par les figures d'Alain, de Clemenceau, de Pierre Mendès France, et, plus tard, par celles de Maurice Faure, René Billères, Michel Crépeau et, bien sûr, de François Abadie François Fortassin était professeur certifié d'histoire-géographie. Né le 2 août 1939 dans cette commune de Sarp, dans la vallée de la Barousse qui lui était si chère, il avait, après des études secondaires au lycée de Saint-Gaudens et des études universitaires à Toulouse, enseigné au lycée Théophile-Gautier, puis au collège Victor-Hugo, à Tarbes. Après quelques engagements syndicaux, sa formation historique, ses convictions républicaines, son attachement à la laïcité et son lien viscéral

l'artisan de la création de la communauté de communes de la vallée de la Barousse. Le défenseur inlassable de son territoire qu'il était s'investit aussi fortement dans le syndicat des eaux de la Barousse et du Comminges. Sa carrière d'élu local conduisit François Fortassin à exercer le mandat de conseiller général du canton de Mauléon-Barousse. Il fut également, durant près de vingt ans, membre du conseil régional de Midi-Pyrénées, où il présida le groupe des radicaux de gauche. D'avril 1992 à mars 2008, il fut président du conseil général des Hautes-Pyrénées, fonction qu'il marqua durablement de son empreinte.

pour soutenir les communes du département. En matière scolaire, le Conseil général réalisa sous son impulsion la réhabilitation de l'ensemble des collèges et soutint le développement d'un pôle universitaire à Tarbes. qui cependant tenait tout particulièrement à coeur à François Fortassin était la reconversion du pic du Midi en un haut lieu touristique, le « vaisseau des étoiles

n'a pas connu la quintessence de la vie et de l'air pur partagé. Je vous en apporte le témoignage, j'étais plus lucide à la montée qu'à la descente François Fortassin n'avait pas prévu de mener cette carrière nationale. Je le cite : « Je ne m'étais pas fixé d'objectif, mais, à un moment donné, François Abadie a vu en moi son successeur. Cela s'est fait comme ça, simplement.

Le Sénat est une chambre de réflexion très utile. Ce que je déplore le plus dans la période actuelle, c'est la dégradation du politique à laquelle on aboutit à travers les réseaux sociaux. Il est bon d'avoir une chambre où peut s'engager la réflexion et qui n'est pas dans la précipitation ou dans l'émotion de l'instant ». Propos à méditer collectivement

sonnaient juste et emportaient bien souvent l'adhésion. Notre collègue était un républicain modéré, mais n'était pas modérément républicain. Il portait au Sénat les valeurs qui étaient les siennes, qu'il s'agisse de la construction européenne - il réclamait inlassablement, même lorsque ce n'était pas du tout la mode, plus d'Europe et mieux d'Europe »-ou de la laïcité, pour laquelle il s'est toujours battu, considérant qu'il fallait affirmer constamment et avec vigueur ces valeurs que la République porte.

J'ai en mémoire ses dernières interventions, à la fin de l'année dernière, sur le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté ou sur deux textes législatifs relatifs aux activités sportives, un autre sujet qui le passionnait. Il déposa encore au début de cette année deux propositions de loi, visant à garantir le principe de l'indépendance de la justice et à rétablir les critères de classement des communes situées en zone de revitalisation rurale. Homme de convictions,

de la tauromachie et celle du rugby, sans oublier, bien sûr, les plaisirs de la table, auxquels l'épicurien jovial qu'il était ne demeurait pas insensible. Je

Oui, François Fortassin a voué l'essentiel de son existence et de son énergie à son travail d'élu et de parlementaire. notre sympathie aux membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen du Sénat et à ses collègues de la commission des affaires sociales. Je voudrais aussi transmettre à chacun des membres de sa famille, ceux qui sont ici présents

le 15 mai dernier, nous avons appris avec une profonde tristesse que François Fortassin venait de nous quitter. Quatre jours plus tard,

Il m'aurait interpellé sur bien des sujets, et, comme il l'a toujours fait, il aurait su faire remonter sa perception du terrain,

conseiller général de 1979 jusqu'en 2015 et président du conseil général de 1992 à mars 2008. En 1982, il a fait son entrée au conseil régional de Midi-Pyrénées ; il y restera

au parti politique qui a toujours été le sien : le parti radical. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le président, les valeurs essentielles du radicalisme s'incarnaient tout à fait dans l'homme qu'était François Fortassin.

il est à l'origine de la création, par son conseil général, du fonds d'aménagement rural et du fonds d'équipement urbain qui permettent de soutenir financièrement les communes du département.

du pic du Midi une priorité à laquelle il est resté attaché jusqu'au bout, et nous sommes nombreux à avoir gravi les pentes du pic du Midi

En cela, il était un sénateur de terrain, pragmatique, libre, loin des dogmes et des postures, respectueux des idées et des convictions des autres. Il était tout simplement un sénateur utile, utile à la fabrique de la loi, utile à la République.

rares étaient les semaines où François Fortassin ne prenait pas l'avion depuis Tarbes ou Pau pour nous rejoindre au Sénat, ce Sénat qu'il aimait tant et qui le lui rendait bien ! Aussi, lorsque depuis plusieurs mois maintenant, ne le voyant plus à notre réunion de groupe, pas davantage dans l'hémicycle ni même au restaurant

je peux dire que François Fortassin fut un vrai, un ardent défenseur des valeurs républicaines. Il y a quelques mois à peine, j'étais j'étais assis à ses côtés dans cet hémicycle lorsqu'il interrogea le garde des sceaux de l'époque sur la nécessité de respecter l'indépendance de l'autorité judiciaire et la séparation des pouvoirs. Cela restera comme sa dernière expression publique au Sénat, elle avait une grande signification. Tous ceux qui l'ont vu à l'oeuvre, en commission comme en séance, gardent de lui le souvenir d'un sénateur profondément attaché aux valeurs de liberté, de solidarité et de tolérance,

Ces valeurs, il les pratiquait au quotidien depuis sa jeunesse, dans l'exercice de ses mandats, mais aussi dans la pratique du sport, plus exactement du rugby et du cyclisme, deux sports parfaitement enracinés, comme lui, dans les Pyrénées.

Qu'il me soit permis aujourd'hui, en ce jour d'étape, à l'approche des Pyrénées, de faire une révélation : si la présence et l'activité en séance publique de François Fortassin durant les chaudes sessions extraordinaires de juillet connaissaient un léger ralentissement, c'était bien sûr parce qu'il ne voulait rien rater des échappées pas plus que des sprints aux arrivées. Il lui arrivait de multiplier les allers et retours entre l'hémicycle et le bureau, tout proche, de son président de groupe et il est bien possible que parfois, un ou deux amendements n'aient pu être défendus

rappelant ainsi avec son bon sens légendaire que « si l'on avait fait manger de l'herbe aux vaches, on n'aurait jamais eu la vache folle. » Cela résume le bon sens, le sens du terrain C'est bien cette voix pragmatique et sincère, celle d'un vrai républicain qui savait toujours ramener les débats à l'essentiel, à savoir l'utilité de la loi, sa perception par les citoyens et ses effets véritables sur le quotidien des Français, oui, c'est cette voix qui s'est tue, cet éclairage qui s'est éteint et qui désormais manquera à tous ses collègues sénateurs. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, homme de passions, homme d'un territoire, homme de son territoire, homme de valeurs fortes, avec la République chevillée au corps, François Fortassin restera une grande figure

ceux qui l'ont connu savent qu'il a désormais trouvé sa place dans ce ciel étoilé des Hautes-Pyrénées, quelque part au-dessus du pic du Midi. Au nom du gouvernement de la République, j'adresse à toute sa famille, à tous ses proches, aux habitants de ce territoire qu'il aimait tant, à ses concitoyens, mes condoléances les plus sincères, et les plus attristées.

avoir remerciés de votre présence nombreuse,

madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le débat relatif au projet de loi visant à rétablir la confiance dans la vie publique est important et fondamental, comme j'ai eu l'occasion de le souligner hier. Les dernières campagnes électorales, les dernières modalités d'exercice du pouvoir, la place des médias dans la vie politique ont mis en exergue l'exaspération, voire le ras-le-bol de nos concitoyens face à la place croissante de l'argent dans la vie politique. Cette question traverse, me semble-t-il, toute la société. Comment ne pas parler de la représentativité des élus ? Comment ne pas parler de la place des médias, de leurs rapports avec puissances d'argent et forces politiques dans un tel débat ?

Si le débat dans sa plénitude n'a pas lieu au Parlement, où aura-t-il lieu ? Au conseil des ministres ? De nombreuses- trop nombreuses ! -irrecevabilités ont été décrétées pour refuser d'emblée l'examen d'amendements, elles au motif que ces derniers n'auraient pas, comme l'exige l'article 45 de la Constitution, de lien direct ou, j'y insiste, indirect avec le projet de loi. Monsieur le président de la commission des lois, vous savez que la réforme constitutionnelle de 2008 avait pour objet d'élargir le droit d'amendement, et non pas de le restreindre. Voulez-vous que je vous donne lecture du rapport de M. Hyest, votre prédécesseur, et de ses interventions en séance publique en la matière ? Vous me direz que c'est le Conseil constitutionnel qui, dans l'un de ces revirements de jurisprudence dont il a le secret, a poussé à restreindre le champ du droit d'amendement. Cela pose une nouvelle fois le problème de la légitimité du Conseil constitutionnel pour décider de l'organisation démocratique de nos institutions. Le Parlement doit défendre ses prérogatives avec fermeté. Le renforcement du pouvoir exécutif décidé et mis en oeuvre très rapidement par M. Macron doit nous faire réfléchir. Le droit d'amendement est crucial pour respecter l'équilibre des pouvoirs et leur séparation. Ce n'est pas au Gouvernement de décider, pour la rédaction de son projet de loi et de ses articles, à cela que revient l'utilisation abusive de l'article 45. Vous donnez au Gouvernement la clef du droit d'amendement, de ce qu'il reste du droit d'amendement. Je vous demande solennellement, monsieur le président de la commission des lois, de revenir sur cette décision, qui met en péril un droit constitutionnel essentiel, lequel caractérise le pouvoir de faire la loi. Acte vous est

je parle sous le contrôle de Mme la garde des sceaux -, une jurisprudence que l'on peut juger sévère, mais qui est en tout cas très nette.

l'a définie la Constitution, celle-ci étant interprétée par le Conseil constitutionnel seul. Notre marge de manoeuvre est, hélas, tout à fait faible dans ce domaine. J'ajoute que ce n'est pas le titre d'un projet de loi qui détermine le champ des amendements possible. Quand il s'agit de parler de confiance ou de moralisation, on pourrait dire que tout se rapporte au projet de loi ; aucune irrecevabilité ne serait alors « recevable »,

déclarés irrecevables le sont réellement, sous réserve de l'appréciation souveraine du Conseil constitutionnel. Si ce texte est adopté, le Conseil constitutionnel peut être amené à statuer sur la régularité de la procédure législative : il dira alors le droit.

que nous voulons réellement nous ancrer dans l'exemplarité et que nous souhaitons une équité entre les élus et eux-mêmes. La bonne intention, c'est bien, mais les Français attendent des actes candidats d'avoir un casier vierge pour ce qui concerne la probité et les atteintes physiques est une attente forte des citoyens, relayée par de nombreuses associations.

Ces sujets troublent le débat politique, ainsi que l'action de milliers d'élus qui travaillent pour l'intérêt général avec abnégation et qui sont pourtant amalgamés avec les affaires d'une poignée d'autres. Nous ne pouvons nous exonérer de ces prises de position à l'heure où nous débattons d'un projet de loi dont l'objet est de rétablir la confiance. En effet, plus de 300 professions exigent un casier vierge pour toute candidature, alors que, aujourd'hui, un candidat à une élection peut

Pourtant, le texte a été adopté par l'Assemblée nationale, et de nombreux experts affirment sa constitutionnalité. Je vous demande donc de penser à l'image que nous donnons de nos hémicycles, à la volonté et à la sincérité que nous nous devons de porter, à la nécessité de prouver nos changements de pratique. Aujourd'hui, ne nous enfermons pas dans les combats de juristes, car ceux-ci sont décalés avec la défiance des citoyens, qui ne voient dans ces querelles que l'envie des élus de ne surtout rien bousculer et ironisent sur le fait que si l'obligation de fournir un casier vierge était votée, il n'y aurait plus de candidat aux élections

Mon amendement vise également à rendre obligatoire la production d'un casier vierge de certaines infractions pour les candidats aux élections municipales, départementales et régionales. Il s'agit du bulletin n° 2,

soigneusement de mentionner les atteintes aux biens, ce qui permet de garantir que des militants politiques s'étant livrés à des actes de désobéissance civile puissent se présenter à des élections. Je pense en particulier aux faucheurs volontaires d'OGM, que je salue, aux actes de résistance contre la ferme des mille vaches ou aux démonteurs des McDonald's, qui luttent contre l'industrialisation à outrance de notre agriculture, ou encore aux actions des « faucheurs de chaises », qui luttent contre l'évasion fiscale. L'amendement

Pour répondre à cette attente, le Gouvernement propose de rendre quasiment automatique le prononcé des peines complémentaires d'inéligibilité lorsqu'un individu est condamné pour avoir commis un crime ou certains délits. De notre point de vue, cette solution n'est pas complètement satisfaisante, puisque, et, d'une certaine manière, à juste titre, le principe d'individualisation des peines fait obstacle à ce que la peine d'inéligibilité soit absolument automatique. Il restera donc toujours possible de passer entre les gouttes. De plus, la solution proposée par le Gouvernement réserve la quasi-automaticité de cette peine complémentaire à une liste limitée de délits, dont on peut contester l'exhaustivité. Enfin, même si, pour ces crimes et délits, le prononcé de l'inéligibilité deviendra la règle et non plus l'exception, il faut souligner que l'avancée attendue est moindre, puisque, à l'heure actuelle, les magistrats disposent déjà de cette possibilité. C'est pourquoi nous proposons de revenir à la proposition adoptée en février dernier par l'Assemblée nationale, qui pose comme préalable à la candidature à une élection le fait de présenter un bulletin n° 2

l'effacement d'une mention sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut se faire à partir d'un délai de six mois après la condamnation.

a fait le choix d'une peine d'inéligibilité obligatoire prononcée explicitement par le juge, en fonction d'une décision spécialement motivée, et qui pourra être écartée expressément en raison des circonstances de l'espèce. Comme la commission, le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

que « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu » notre amendement tend à respecter aussi bien la liberté de l'électeur que l'indépendance de l'élu, dans la mesure où il ne vise que des comportements malhonnêtes ayant été prouvés et condamnés lors de procès réguliers et contradictoires. En outre,

Enfin, si ces dispositions demeurent punitives aux yeux de certains, il faut rappeler que la jurisprudence constitutionnelle, que, madame la garde des sceaux, vous ne pouvez ignorer, a évolué depuis la censure de l'article 7 du code électoral, de sorte qu'il n'existe pas d'interdiction de principe des peines obligatoires. Dans sa jurisprudence la plus récente, que vous connaissez très bien, le Conseil constitutionnel subordonne leur conformité au principe d'individualisation des peines en se fondant sur un certain nombre de critères, que remplit la condition d'éligibilité. En conséquence, si l'inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire est de droit, elle n'est pas automatique, le juge pouvant à tout moment ordonner son omission.

Nous connaissons tous le cas de ce maire, dont j'aurai la délicatesse de ne pas nommer la commune, qui, condamné pour agression sexuelle à l'égard de l'une de ses employés, a néanmoins échappé à une peine d'inéligibilité et continue tranquillement d'exercer ses fonctions, alors que sa victime, elle, est complètement détruite et ne peut plus travailler.

projet de loi réserve le nouveau régime de peines complémentaires d'inéligibilité aux crimes, ainsi qu'à une liste de délits. Or le problème des listes, c'est qu'elles sont rarement exhaustives. S'agissant des infractions susceptibles d'entraîner ces nouvelles peines d'inéligibilité, on peut s'étonner que les rédacteurs de l'article aient considéré que les délits financiers justifient un traitement spécial, mais oublié les atteintes aux personnes. Il Il serait curieux de supposer que les Français n'entendent pas être représentés par des individus de petite probité, mais qu'ils acceptent de l'être par des personnes condamnées pour violences, harcèlement sexuel ou moral

L'élargissement de la liste des infractions concernées ne doit pas, de mon point de vue, susciter une extension difficilement contrôlable de celle-ci. Or l'ajout à cette liste du délit de harcèlement conduirait nécessairement

Je ne résiste pas à la tentation de souligner cette attention toute particulière du Gouvernement pour la délinquance financière.

portait sur la version antérieure de l'amendement de M. Collombat, qui a été rectifié pour ne plus viser que l'escroquerie en bande organisée. Je me demande si votre objection ne tombe pas compte tenu de l'effort de précision accompli par notre collègue. Il s'agit tout simplement de considérer que les délits entachant la probité dans la gestion des deniers

des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Il constitue un délit d'appropriation illégitime, voisin de l'abus de confiance. Ainsi, l'abus de biens sociaux est à l'exact opposé de la mission de l'élu. Il représente un manquement grave aux responsabilités dont il a la charge.

Mme la garde des sceaux. Je propose un amendement visant à la suppression de l'article 1 qui modifie le délit de prise illégale d'intérêts. La commission des lois du Sénat a adopté un amendement tendant à modifier la définition du délit de prise illégale d'intérêts, au motif que la jurisprudence retiendrait une acception trop imprécise de la notion d'intérêt, permettant notamment de sanctionner la prise d'un intérêt moral, voire une simple erreur de forme. Il en résulterait pour les élus locaux une forte exposition à un risque de condamnation pénale pour des manquements purement formels. Le Gouvernement conteste une telle analyse et souhaite maintenir ce texte dans sa rédaction actuelle. La prise illégale d'intérêts vise à s'assurer que le jugement des décideurs publics ne soit pas altéré par un autre intérêt que l'intérêt général, d'une part, et que ces décideurs ne puissent pas être suspectés de complaisance dans l'exercice de leurs prérogatives, d'autre part. Cela permet ainsi de sanctionner des personnes dépositaires de l'autorité publique

Il convient enfin de souligner que les juridictions font une application particulièrement limitée de ces dispositions, dans la mesure où le nombre de condamnations annuelles pour des faits de prise illégale d'intérêts oscille autour d'une quarantaine Une modification de l'incrimination n'aurait donc d'autre effet que de faire diminuer encore davantage le nombre de ces condamnations. C'est pourquoi l'article 1 doit être supprimé.

d'élus dont les comportements ne portaient pourtant nullement atteinte ni à la probité ni même à l'objectivité, mais qui avaient pris part à des délibérations

cette rédaction équilibrée consistant à définir l'intérêt qui caractérise la prise illégale d'intérêts comme « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général

a représenté une des avancées les plus significatives du droit au cours de ces dernières années. Instrument essentiel de la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance financière, le parquet national financier demeure cependant confronté à un problème, celui qui est posé par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, qui fait de la commission des infractions fiscales- organisme placé auprès du ministre de l'économie et des finances, le « juge d'instruction » des affaires de fraude pouvant donner lieu à une transmission au pénal. C'est ce que l'on appelle familièrement le « verrou de Bercy Il importe que cette exclusive à la nécessaire prolongation de l'investigation lancée dans le cadre d'autres contrôles ou enquêtes soit levée, afin que les administrations ou les services qui, dans leurs activités courantes, auraient repéré une situation constitutive d'une fraude fiscale avérée puissent engager les poursuites nécessaires, quitte à mettre en oeuvre des mesures conservatoires, comme la saisie de sommes en transit illégalement, par exemple, et à aviser l'administration fiscale au plus haut niveau du produit de leurs investigations. Cette question a notamment été soulevée par un mémorandum remis en référé par le Premier président de la Cour des comptes au Premier ministre en août 2013. Ce document souligne la nécessité d'un renforcement de la coopération entre la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects. par souci d'égalité des citoyens devant la justice et devant l'impôt, le « verrou de Bercy », système donnant à l'administration fiscale la main sur les poursuites pénales en matière fiscale, doit, selon nous et beaucoup d'autres, être supprimé.

qu'elles ne garantissent pas la victoire au bout et qu'il vaut mieux utiliser cette arme pour faire pression sur les fraudeurs, afin de récupérer un peu d'argent dans les caisses de la République ...

contre la fraude, notamment quand celle-ci est révélée de manière incidente dans le cadre d'autres infractions. Il est anormal que l'accès à la justice soit conditionné à l'avis d'une administration

2016, le Sénat a voté la demande de levée du « verrou de Bercy

C'est une question de morale, une question de vertu, comme on le dit dans notre République, mais c'est aussi une question d'efficacité. En effet, vous le savez, pour que l'administration fiscale puisse transmettre un dossier à la justice,

de la commission des finances que de la commission des lois, si bien que je suis naturellement embarrassé de ne pas pouvoir me prononcer de manière éclairée sur cette question.

au fraudeur mais de lui faire rendre l'argent, ce qui n'est pas la même chose ! La responsabilité principale des poursuites ou de la négociation destinée à obtenir un maximum de retours cadre du dialogue entre le contribuable fraudeur et l'administration relève donc du ministère des finances. En somme, ceux qui ont inventé le « verrou de Bercy » l'ont fait dans l'intérêt de l'État et la loi

naturellement instruite dans des conditions tout à fait ordinaires. Pour toutes ces raisons, et dans le souci de ne pas improviser une réponse qui ne serait pas élaborée avec l'accord de la commission des finances,

qui vise à autoriser l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, soit sans plainte de l'administration fiscale ni saisine de la commission des infractions fiscales, soit sur plainte de l'administration mais sans saisine

que la pratique de l'administration fiscale n'est pas guidée par le principe d'égalité devant la loi, lorsqu'elle effectue des contrôles et lorsqu'elle dépose plainte pour fraude fiscale. Or le Gouvernement ne partage évidemment pas ce soupçon.

De toute façon, la correctionnalisation potentielle de l'ensemble des fraudes fiscales connexes à d'autres infractions sur l'initiative des seuls parquets entraînerait également la nécessité de définir une politique pénale, de de manière à ne pas « surpénaliser » la fraude fiscale et à traiter de manière égalitaire les citoyens dans toutes les juridictions de France. Je dois en effet souligner que, dans la majorité des cas, l'application des pénalités fiscales exclusives de bonne foi suffit à réparer le préjudice financier subi par le trésor public et, plus généralement,

Le Gouvernement ne souhaite donc pas généraliser la sanction pour fraude fiscale par le juge pénal à tous les cas de fraude. Cela paraîtrait totalement disproportionné et ne serait pas conforme au cadre constitutionnel de la lutte contre la fraude. La saisine de la commission des infractions fiscales contribue à avoir une vision nationale et homogène, qui permet de justifier le dépôt de plaintes pour fraude

Parler de « surpénalisation » de la fraude fiscale ne manque évidemment pas de sel

cas presque semblables ne sont pas nécessairement traités avec la même équité ou la même approche. Sur ce point, il faudra une évolution si

participerait de la démarche volontariste de lutte contre l'évasion fiscale.

Par cet amendement, nous proposons d'associer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux dispositions sur la prévention des conflits d'intérêts

d'intérêts. Ils ont conduit le bureau du Sénat, dès 2011, à mettre en place un dispositif interne de déclarations d'activités et d'intérêts des sénatrices et des sénateurs. Ont également été formulées des propositions ayant inspiré le dispositif de prévention et de traitement des conflits d'intérêts, qui va jusqu'à conférer au bureau un pouvoir de sanction disciplinaire envers les membres du Sénat qui n'auraient pas respecté leurs obligations déontologiques en la matière. Pour autant, il nous semble nécessaire d'aller plus loin et, surtout, de sortir des murs et de l'entre-soi.

avec l'administration fiscale -et publier les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts de certains élus, membres du Gouvernement, collaborateurs et dirigeants d'organismes publics. Elle peut également être consultée par des élus qui seraient confrontés, dans l'exercice de leurs fonctions, à des questions de la vie publique participe en amont à la détermination des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires. L'expérience acquise et son statut indépendant

relative à la transparence de la vie publique, qui évoquait « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés ». Dans un souci de clarté juridique, il est préférable que cette même définition soit retenue afin, bien sûr, d'éviter une démultiplication inutile des définitions.

Je ne résiste pas à la tentation de féliciter le Gouvernement d'avoir modifié la définition

loin s'agissant de conflits possibles entre intérêts publics et intérêts publics aboutirait à des contradictions perpétuelles. Nous sommes tous les élus d'un département. au Parlement, nous défendons telle entreprise qui est en difficulté dans ce département, tel service public que nous voulons soutenir, tel aménagement nécessaire, on on pourra arguer que nous utilisons notre mandat national pour défendre un intérêt local. Mais nous sommes les élus de la République, les élus de l'ensemble des collectivités et des citoyens, et il nous appartient effectivement

amendements présentés, et je le dis avec le sens de l'euphémisme auquel je suis attaché.

Il s'agit donc pour moi non pas de les remettre en cause, mais, au contraire, d'en garantir le bon fonctionnement, de renforcer leur pouvoir et de les valoriser. Pour ce faire, nous devons les protéger contre toute dérive possible, notamment en termes de conflit d'intérêts. C'est le sens de ces deux amendements, qui tendent à renforcer les règles des assemblées relatives à la composition et au fonctionnement des groupes interparlementaires d'amitié, en prévoyant que ces assemblées adoptent un corpus de règles destinées spécifiquement à prévenir

n° 226 rectifié tend à prévoir que chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles les parlementaires souhaitant devenir membres d'un groupe interparlementaire d'amitié déclarent les intérêts qu'ils détiennent dans les pays

à la consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire afin de définir les règles destinées à prévenir les conflits d'intérêts. Au travers de ces deux dispositifs, il s'agit de renforcer le rôle des parlementaires dans leur fonction, en mettant en place un garde-fou contre des dérives

dans la loi des dispositions relevant de l'autonomie de chacune de nos assemblées. J'ajoute que la disposition qui imposerait à un membre du Parlement ayant de la famille à l'étranger

La séance est reprise.

le Premier ministre irakien, Haïder Al-Abadi, a annoncé la libération de Mossoul, l'ancienne Ninive, berceau des civilisations assyrienne et chaldéenne, qui a brillé de tant de feux et a donc suscité tant de convoitises. Cette victoire est le fruit de la détermination des forces irakiennes et des peshmergas kurdes, qui, ensemble, en première ligne, ont subi des milliers de pertes pour se réapproprier les rives du Tigre. est aussi le fruit de l'engagement, sans faille, des forces de la coalition internationale, dont la France, auprès des Irakiens. La libération de Mossoul porte un coup, que nous espérons fatal, à l'État islamique et à sa folie destructrice. Saluons ici cette victoire comme le signal de la reconstruction de l'Irak et d'un Moyen-Orient qui a soif de paix et de stabilité. Mossoul est libérée du joug de l'État islamique ; mais Mossoul n'est qu'un champ de ruines, et sa population sort de l'enfer. Aujourd'hui, des questions essentielles se posent : comment sauver ces vies hagardes, ces familles brisées, ces quartiers en lambeaux ? Comment réenclencher la vie ? Comment réenclencher l'économie ? La coalition a-t-elle réfléchi au volet humanitaire ? Une autre question a trait à la position de la France. La reconquête de Raqqa, l'autre capitale des forces obscurantistes, semble en bonne voie, sa future libération dessine un horizon nouveau pour la Syrie. À cet égard, je salue nos forces armées, leur expertise, leur dévouement et leur professionnalisme. N'y a-t-il pas là, en Irak et en Syrie, une opportunité pour relancer un processus politique régional aujourd'hui complètement enlisé ? Comment la France,

: la libération de Mossoul, grâce à la reconquête, par les forces irakiennes et celles de la coalition, de cette ville qui était occupée par les djihadistes depuis que ceux-ci y avaient annoncé la proclamation d'un prétendu khalifat à l'été 2014.

coalition au sein de laquelle la France a joué un rôle majeur. Je rappelle que nous avons appuyé les forces irakiennes grâce à notre aviation, basée en Jordanie et aux Émirats arabes unis, et grâce à nos pièces d'artillerie, déployées en périphérie de Mossoul. Nous leur avons également fourni du matériel et des renseignements. Enfin, nous avons contribué à la formation d'un certain nombre d'unités, grâce à des instructeurs déployés à Bagdad et à Erbil. Je souhaite, moi aussi, rendre un vibrant hommage aux forces françaises, à tous ces militaires déployés au Levant, qui ont pris une part active à cette reconquête. Néanmoins, il reste beaucoup à faire. C'est sûr ! La victoire finale n'est pas encore toute proche. Daech continue de contrôler un certain nombre de territoires, en Irak comme en Syrie.

que la reconquête ne sera pas seulement militaire : un processus politique et un accompagnement économique devront être organisés, sous l'égide de la coalition dont la France fait partie. La parole

Vous souhaitez lui donner une autre orientation, le financement des grands projets d'infrastructures, que vous chiffrez à 10 milliards d'euros, afin que les poids lourds circulant sur nos routes contribuent davantage à l'entretien et, surtout, à la modernisation des différents axes stratégiques de notre pays. Parmi les pistes de réflexion, vous évoquez l'expérimentation de ce dispositif dans des régions volontaires ; la mise en place de péages sur certaines sections de routes nationales, afin de ne pas pénaliser les transports de proximité ; ou encore la création d'une taxe spécifique dédiée aux besoins en équipement. Comme beaucoup, je soutiens cette proposition, qui permettrait, d'une part, de financer l'entretien et l'aménagement de notre vaste réseau routier et, d'autre part, de soulager les collectivités propriétaires, qui aujourd'hui ont du mal à assumer ces missions.

Je songe à l'état de nos réseaux de transports, qui se dégrade, ainsi qu'à la qualité de l'environnement, notamment- vous l'avez souligné -dans les villes et les villages traversés par ces infrastructures.

pu recourir, principalement pour les poids lourds étrangers. L'objectif est bien de dégager de nouvelles ressources tout en encourageant les comportements les plus vertueux au regard de l'environnement. Tous ces points seront inscrits à l'ordre du jour des assises de la mobilité, qui se tiendront à partir de septembre prochain.

Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Ah ! Alors que certaines de vos promesses en faveur du pouvoir d'achat ont disparu- je pense à la défiscalisation des heures supplémentaires -, vous donnez la priorité à la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des Français. C'est une très bonne chose ! Après de nombreuses hésitations et de nombreux revirements, il a été précisé hier que cette mesure entrerait en vigueur progressivement dès l'année prochaine.

Je vous pose la question : si cette taxe est injuste, où se trouve la justice pour les 20 % de Français qui continueront de la payer et pour nos concitoyens assujettis à la taxe foncière, laquelle est assise sur les mêmes valeurs locatives ? Certes, le calcul de la taxe d'habitation souffre aujourd'hui d'une certaine obsolescence, en raison de l'absence d'actualisation des valeurs cadastrales depuis 1970 et de l'existence de taux d'imposition très différents selon les communes. Ces taux sont d'ailleurs parfois plus élevés dans des zones rurales ou urbaines défavorisées qu'à Paris par exemple. la solution n'est-elle pas plutôt d'assurer une réforme structurelle, visant à rendre cet impôt plus juste, plutôt que d'en exonérer seulement une partie des Français, au détriment des finances des communes ?

La parole est à M. Philippe Esnol, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen.

Une telle concertation est en effet attendue par les élus, attachés à la libre administration des collectivités territoriales et à son corollaire, leur autonomie financière. Elle se révèle par ailleurs indispensable pour trouver, à terme, des recettes pérennes pour les collectivités, plus que des compensations qui- les expériences passées l'ont prouvé malheureusement -n'ont jamais vocation à durer. M. le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a même eu l'occasion, dans la foulée, de préciser en réponse à une question de notre collègue Bernard Delcros que les maires pouvaient être rassurés dans la mesure où vous saviez tous deux, par expérience, que la taxe d'habitation constituait une recette majeure des collectivités territoriales.

Ainsi, même si cet impôt est injuste pour les contribuables comme pour les territoires, en raison de valeurs locatives cadastrales obsolètes et des inégalités de richesses entre communes, et s'il est, en conséquence, souhaitable de le réformer, notre devoir est de veiller à ce que cela ne soit pas mené au détriment des collectivités. Je rappelle que ces dernières ont, en outre, déjà largement pris leur part au redressement des comptes publics ces dernières années. C'est pourquoi, alors qu'a été réaffirmée hier la mise en oeuvre dès 2018 de votre engagement d'exonérer 80 % des ménages de la taxe d'habitation, je souhaiterais vous poser deux questions. D'une part, quelles sont les mesures de compensation envisagées permettant de tenir votre engagement de « prévisibilité » et de donner aux communes des garanties de l'État à long terme ? D'autre part, comment comptez-vous associer les premiers concernés, à savoir les élus locaux, qui s'interrogent, en pareilles conditions, quant à leur capacité à financer nos services publics de proximité, essentiels et plébiscités par les Français, tout en maintenant l'équilibre de leur budget ? Il était prévu d'ouvrir ce qui n'était hier encore qu'un chantier lors de la conférence des territoires programmée lundi. Pouvez-vous aujourd'hui nous en préciser les modalités ? La parole est à M. le ministre

en marche. Monsieur le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, « l'Europe est en passe d'atteindre ses objectifs pour 2020 en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique et la production d'énergie de sources renouvelables Telle est la conclusion rassurante du dernier rapport publié par la Commission européenne. Ce constat encourageant ne doit pourtant pas masquer les difficultés rencontrées dans l'adaptation du système énergétique européen à la lutte contre le changement climatique. Malgré les objectifs ambitieux de la loi de transition énergétique, la France atteindra difficilement sa cible de 23 % d'énergies renouvelables en 2020. Quant à l'Allemagne, non seulement elle ne parviendra probablement pas à réduire d'ici là, comme annoncé, ses émissions de CO2 de 40 %, mais son gouvernement a récemment repoussé à 2040 la sortie du charbon. Dans ce contexte, il est important d'accélérer et d'encourager l'innovation pour une riposte mondiale à long terme face au changement climatique. énergétique visant à ramener à 50 % la part du nucléaire dans la production d'électricité à l'horizon 2025, vous avez annoncé hier vouloir fermer jusqu'à dix-sept réacteurs. Toutefois, un important programme de rénovation du parc nucléaire français doit permettre d'allonger la durée de vie des centrales et de susciter des retombées importantes pour nos entreprises. Monsieur le ministre d'État, quelle est votre vision du mix énergétique dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Allez-vous préserver la complémentarité des énergies de base, nucléaire et hydrocarbures, qui satisfont encore la majorité de la consommation d'énergie, d'une part, et des énergies renouvelables, d'autre part ? Il faudra aussi trouver un équilibre entre innovation et précaution et éviter tout attentisme pour moderniser l'économie et prendre la direction de la lutte contre le réchauffement climatique.

ce dont nous avons besoin, d'abord, c'est d'un débat serein, et j'ai souhaité hier que nous ouvrions ce débat. Ce dernier doit être cohérent et transparent,

avec l'horizon qui a été fixé, et que vous avez rappelé, par la loi de transition énergétique. Ce texte est particulièrement ambitieux : croyez-moi, j'en ai bien conscience. Dans cette loi, entre autres objectifs,

portée au potentiel de toutes les énergies : nous devons tout faire pour accélérer le développement des énergies renouvelables et retrouver notre souveraineté de choix en matière énergétique. La programmation pluriannuelle de l'énergie se fera dans un dialogue renforcé avec tous les acteurs, syndicats, industriels, associations,

injuste, certes, mais dont les valeurs de référence commençaient justement à peine d'être révisées, notamment l'allégement de la fiscalité pesant sur les logements locatifs sociaux, la taxe d'habitation va donc être réformée. Nul doute que les contribuables qui ne la paieront plus du tout seront, dans un premier temps, satisfaits. Mais il est clair, vu les autres mesures annoncées, qu'il s'agit là de faire passer la pilule amère de la hausse de la CSG et celle de l'absence de coup de pouce pour le SMIC, en attendant la hausse des taxes sur l'essence, le tabac et le maintien d'une TVA à 21,2 %. Cette annonce masque également et surtout l'indécence de l'exonération de l'ISF pour les fortunes mobilières. Eh oui ! D'un côté, 3 milliards d'euros à partager entre 28 millions de redevables

comment allez-vous assurer aux collectivités locales, et notamment aux communes, dont la taxe d'habitation conditionne l'autonomie financière, les ressources que cette réforme risque de leur faire perdre ? Ne serait-il pas préférable de prolonger et de renforcer les actuels abattements et dégrèvements applicables à la taxe d'habitation afin de limiter l'effort fiscal des redevables ?

villes et des campagnes. Ces derniers ne sont toujours pas invités à participer lundi à cette grande conférence nationale des territoires : ne nous donnez pas de leçons en matière de consultation, nous subissons aujourd'hui les choix politiques que vous nous imposez

juillet dernier, vous avez assuré publiquement qu'une solution n'était pas loin dans le dossier de reprise de l'équipementier automobile creusois GM&S Industry. Ce dernier est actuellement en liquidation judiciaire, avec poursuite de l'activité jusqu'au 19 juillet prochain. Dans votre communiqué en date du 21 mai dernier, vous sembliez déjà confiant quant aux propositions faites par les deux donneurs d'ordre, PSA et Renault, au sujet de l'augmentation du volume des commandes. Or la confirmation précise et assurée de ces engagements se fait toujours attendre. La disparition de cette société représenterait un choc économique et social dramatique pour La Souterraine, cité de 5 000 habitants, et affecterait fortement tout un bassin de vie, à cheval sur trois départements. Je souhaite que votre optimisme enthousiaste se concrétise, afin d'en finir avec une histoire récente douloureuse, marquée par trois redressements judiciaires en moins de huit ans et de nombreux engagements non tenus, d'où l'épuisement des salariés et des réactions virulentes, traduction de leur colère et de leur désespoir. Cette stratégie de rapport de forces a permis de mettre à l'ordre du jour des discussions des points essentiels. À quel stade en sont ces discussions ? Aujourd'hui même, une rencontre, qualifiée par beaucoup de « réunion de la dernière chance », et à laquelle les deux sénateurs du département n'ont pas été conviés, se tient à Bercy. Nous ne pourrons nous satisfaire d'une demi-solution génératrice, à moyen terme, de nouvelles exaspérations. Enfin, je veux saluer ici la mobilisation de la région Nouvelle-Aquitaine dans ce dossier très difficile, notamment pour le soutien à toutes formes de diversification, mais également l'implication de l'État au cours de ces derniers mois : financement de l'activité partielle, CICE, non-exigibilité de la dette sociale et fiscale. Ces efforts, accompagnés par les élus et la population locale, ne sauraient rester vains, la qualité du savoir-faire de cette entreprise étant reconnue de tout le secteur automobile. Que fait l'État pour contribuer à un avenir crédible et pérenne pour ce site industriel ? Quelle sortie de crise attend ses 277 salariés, leurs familles et leur territoire ?

donc pas nécessaire de rappeler la mobilisation de tous les acteurs et du Gouvernement pour trouver, dans un esprit de dialogue constructif, l'issue la plus favorable possible, dont nous savons qu'elle ne pourra pas concerner l'ensemble des salariés, et les solutions permettant de sortir de cette situation. Il faut d'ailleurs saluer l'esprit de responsabilité des salariés et de leurs représentants en vue de contribuer à la recherche d'une meilleure solution. Même s'il y a eu des moments de colère, il était nécessaire de raison garder ; ils ont en ont fait la démonstration. C'est ainsi que nous trouverons les solutions pour La Souterraine, ce territoire

en volume et en chiffre d'affaires. Nous avons déjà obtenu un renfort important de ces engagements, à hauteur de 22 millions d'euros, de la part des deux principaux clients, Peugeot et Renault. Il faut également obtenir du repreneur des engagements d'investissement

à Montpellier, un conseil de métropole extraordinaire était convoqué. Son ordre du jour martial comprenait la destitution, puis le remplacement de sept vice-présidents. Ces vice-présidents, six maires et un premier adjoint-l'un d'entre eux avait démissionné afin de ne pas être exécuté -, de toutes les sensibilités politiques, représentaient les principales villes de notre intercommunalité. Ces élus de qualité, d'expérience, ont été démis de leurs fonctions au seul motif qu'ils ont refusé de s'inscrire au groupe En Marche constitué par le président de notre métropole. Cette condition était préalable au maintien de tous les vice-présidents et au choix des remplaçants de ceux qui refusaient. La population et les élus découvrent, horrifiés, ces méthodes politiques d'un autre temps, et un doute perceptible s'installe sur le nouveau parti politique La Ces interrogations se renforcent, dès lors que le président de la métropole affirme publiquement, et à tout propos, bénéficier de l'encouragement et du soutien du chef de l'État. Mes convictions gaullistes, ma conception de l'intercommunalité, selon laquelle nous représentons nos villes et non un parti politique, font que je n'accepterai jamais cette remise en cause cynique de la démocratie locale et de l'esprit des lois de décentralisation. Je veux croire qu'il ne s'agit là que d'un cas isolé, de la dérive d'un seul homme et de l'usurpation d'un soutien inconditionnel des responsables de l'État. La confiance dans la vie politique, dont nous débattons actuellement au Sénat, impose aux élus le respect de la probité et de la démocratie ; pas l'une sans l'autre Ces règles s'appliquent sur tout le territoire et dans toutes les institutions gérées par des élus. Cette affaire est suffisamment grave, monsieur le Premier ministre, pour que le Gouvernement rassure le Sénat sur sa volonté de faire respecter partout les valeurs de la République.

l'exécutif de la métropole a été partiellement renouvelé. Comme vous le savez, le code général des collectivités territoriales fixe un certain nombre de règles entourant la délégation de fonctions par le président à des vice-présidents au sein des métropoles. Le code et la jurisprudence encadrent également les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être retirées et les circonstances dans lesquelles le conseil communautaire est appelé à en connaître. Au-delà des dispositions législatives et réglementaires, la composition des exécutifs s'efforce, en règle générale, de refléter la pluralité des communes membres, gage d'un fonctionnement harmonieux des métropoles, auquel le Gouvernement ne peut qu'être attaché, à Montpellier comme ailleurs. Cependant, il n'appartient pas au Gouvernement de se prononcer en opportunité s'agissant du respect des équilibres qui relève de l'appréciation de chaque collectivité, qu'elle soit de droit commun, comme la métropole de Montpellier, ou à statut particulier. Vous le savez- et ce n'est pas ici que l'on me démentira -, la libre administration des collectivités territoriales est un principe consacré par la Constitution en son article 72, alinéa 3. Je sais combien la la Haute Assemblée veille, en toutes circonstances, au respect strict de ce principe constitutionnel ; il n'appartient donc pas au Gouvernement de se prononcer

Depuis le 1 juillet et l'inauguration de deux lignes à grande vitesse, Rennes n'est plus qu'à 1 heure 25 de Paris et Bordeaux à 2 Mais, lors des festivités en gare de Bordeaux, les silences et les déclarations ambiguës des membres du Gouvernement concernant le prolongement de la LGV jusqu'à Toulouse ont jeté un trouble, pour ne pas dire un froid. Monsieur le Premier ministre, alors qu'en mars 2015 la commission d'enquête avait émis un avis négatif pour les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, six mois plus tard, le Gouvernement de l'époque s'était engagé à poursuivre ces projets. De fait, le 5 juin 2016, était signé le décret déclarant d'utilité publique la réalisation de ces deux LGV. Le 28 juin dernier, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de la déclaration d'utilité publique- DUP -des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, en s'appuyant, pour l'essentiel, sur l'absence de solidité financière. Or, vous le savez, un comité de financeurs, auquel participent toutes les collectivités locales de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie concernées par le projet, a été lancé il y a un an pour répondre à cet enjeu. Un cabinet indépendant, mandaté par ces collectivités, fera d'ailleurs prochainement des propositions innovantes, réalistes et concrètes de financement. Tant et si bien que le motif d'annulation de cette DUP ne devrait plus avoir de raison d'être. Monsieur le Premier ministre, comment peut-on imaginer que la région Occitanie et la métropole toulousaine, première métropole de France en termes de croissance démographique et économique, ne soient pas intégrées au réseau ferroviaire à grande vitesse ? Lors de la campagne présidentielle, M. Emmanuel Macron avait d'ailleurs réaffirmé « son complet soutien » à la LGV Bordeaux-Toulouse. je vous demande, monsieur le Premier ministre, de bien vouloir me confirmer aujourd'hui la volonté de l'État de poursuivre la réalisation de ces deux LGV.

par le tribunal administratif de l'une des trois déclarations d'utilité publique nécessaires pour la réalisation de ce projet. Depuis le 1juillet dernier, Bordeaux n'est plus qu'à 2 heures de Paris et Toulouse à 4 heures 10, mais je mesure les attentes des Toulousaines et des Toulousains. Néanmoins, la branche Bordeaux-Toulouse nécessite de mobiliser encore 6 milliards d'euros. Oh là là ! Or personne ne peut plus ignorer l'impasse dans laquelle l'addition des engagements pris au cas par cas nous a placés il manque aujourd'hui 10 milliards d'euros pour assurer la pérennité de nos réseaux et honorer les engagements pris par les précédents gouvernements, dont 7 milliards d'euros pour les seules nouvelles infrastructures. C'est dans ce contexte que le Président de la République a, dans son discours de Rennes, annoncé une pause. Cette pause doit permettre de définir le chemin par lequel nous allons répondre au mieux aux besoins de transport des habitants de la région, et rechercher une trajectoire soutenable en termes de financement de ce projet. Ce chemin sera à tracer dans un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs concernés par cet ambitieux projet : les citoyens, les élus, les associations, les entreprises. Je sors d'une réunion avec le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et je rencontrerai, dans les tout prochains jours, la présidente du conseil régional d'Occitanie pour échanger sur ce projet. Je ne doute pas que nous arrivions, ensemble, à trouver des solutions soutenables pour ces projets.

socialiste et républicain. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre, et j'y associe mes collègues du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise, particulièrement Laurence Rossignol, Dominique Bailly, Jean-Claude Leroy et Christian Manable. La réponse de Mme la ministre des transports à la question relative au calendrier de réalisation du projet du canal Seine Nord, posée par notre collègue Jean-François Rapin, a véritablement jeté un « pavé dans le canal Seine Nord Nous entendons la réponse de Mme la ministre concernant l'attente d'une loi de programmation quinquennale, mais celle-ci ne peut concerner le canal Seine Nord, projet structurant pour notre région Hauts-de-France, pour notre territoire national ainsi que pour le territoire Nord Europe. Le projet de canal Seine Nord connaît une relance en 2007-2008, lors du Grenelle de l'environnement. Un rapport, commandé en 2012, en évalue les problématiques écologiques et de financement. En avril 2013, une mission présidée par le député-maire Rémi Pauvros reconfigure le projet, y compris sur son aspect budgétaire. En 2015, l'Union européenne annonce une contribution à hauteur de 42 %, soit 1,8 milliard d'euros. Les acteurs institutionnels, tous engagements partisans confondus, se sont engagés budgétairement à démarrer les travaux à la fin 2017. Un accord a été conclu entre l'État et les régions Île-de-France et Hauts-de-France ainsi qu'avec, notamment, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise. Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, alors premier vice-président du conseil régional Hauts-de-France délégué aux transports et aux infrastructures de transport, plaidait également pour un démarrage rapide des travaux. Enfin, en mars 2017, le Président de la République, alors candidat, déclarait : « Je confirme les trois grands projets en cours dont les déclarations d'intérêt public sont en train d'être obtenues, c'est-à-dire le Bordeaux-Toulouse, le Lyon-Turin et le canal Seine Nord qui sont trois gros travaux d'infrastructure ». Pour des raisons économiques, sociales et environnementales, la réalisation de ce projet ne peut plus attendre. Monsieur le Premier ministre, le Gouvernement doit passer à l'action.

Je sais leur attachement à ce projet et les attentes qu'il a fait naître. Votre question en témoigne et me donne l'occasion de préciser de nouveau la démarche engagée par le Gouvernement. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer devant votre Haute Assemblée, des engagements ont été pris sans vision d'ensemble, qui représentent une impasse de 10 milliards d'euros sur le quinquennat. Il n'est plus possible de promettre de manière irresponsable des projets pour lesquels l'État ne dispose pas aujourd'hui des ressources nécessaires. Les assises de la mobilité seront lancées à l'automne et permettront d'associer l'ensemble des acteurs concernés, citoyens, collectivités, associations et entreprises. Il s'agira de conduire un travail d'identification des besoins de chaque territoire. Il s'agira également de réfléchir aux ressources qui peuvent être mobilisées. Il s'agira, enfin, de disposer d'une vision d'ensemble pour répondre à un impératif, celui d'adapter les besoins et les ressources. Cette approche ne peut qu'être partagée par le Sénat, si j'en crois les nombreux rapports publiés depuis quelques mois par vos commissions. Nous serons à l'écoute des collectivités et des élus tout au long du processus. Le Sénat y sera, naturellement, pleinement associé dès le lancement des assises et jusqu'à la présentation du projet de loi de programmation, qui nous permettra de trouver ensemble des réponses concrètes aux besoins de mobilité de nos territoires, soutenables financièrement.

et en application de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, M. le Premier ministre, par lettre en date du 11 juillet 2017, a demandé à M. le Président du Sénat de lui faire connaître l'avis de la commission du Sénat compétente en matière d'activités financières sur le projet de nomination de M. Robert Ophèle aux fonctions de président de l'Autorité des marchés financiers. Cette demande d'avis a été transmise à la commission des finances. Acte est donné de cette communication. Nous reprenons la discussion du projet de loi,

détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en oeuvre. » Cet amendement tend à prévoir la nomination d'un déontologue, afin d'apporter le regard d'un spécialiste de la déontologie parlementaire.

un grand nombre de nos concitoyens se sont étonnés que les règles de déontologie relevant de chaque assemblée soient déterminées et appliquées par les parlementaires eux-mêmes. Nous sommes tous en la matière juges et parties. Cet amendement vise donc à réintroduire un conseil extérieur sur ces questions, à travers l'accompagnement d'un déontologue professionnel. Quel Quel est l'avis de la commission ? L'avis est défavorable. Le comité de déontologie du Sénat est remarquablement présidé par un de nos collègues qui a toutes les qualités requises, notamment en termes d'indépendance et d'élévation morale, pour assumer cette fonction.

un parlementaire à faire cesser immédiatement la situation de conflit d'intérêts dans laquelle il peut se trouver revient à nier son autonomie d'appréciation sur le point de savoir s'il y a, ou non,

Mme Sylvie Robert. L'amendement tend à prévoir un dispositif normatif dans l'hypothèse où un parlementaire demeurerait en situation de conflit d'intérêts. En l'état, le texte est muet sur cette éventualité. Ainsi, le comité de déontologie de chaque assemblée pourrait saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu'il constate des irrégularités en la matière.

permet pas de porter ce genre d'appréciation. Par ailleurs, il appartient au bureau de chaque assemblée, en raison du principe d'autonomie des assemblées parlementaires, après avoir obtenu l'appui du comité de déontologie parlementaire, de mettre en oeuvre les procédures très précises et efficaces qui sont prévues par notre réglementation interne, et que j'ai d'ailleurs rappelées dans mon rapport. On ne voit pas quelle portée pourrait avoir cet amendement dès lors que la HATVP ne pourrait pas agir dans ce domaine d'une manière pertinente. Nous considérons également qu'il appartient aux assemblées de prévoir les sanctions appropriées en cas de manquement à une règle relative aux conflits d'intérêts. Je mets aux voix

cela ne m'est encore jamais arrivé ! Toutefois, si les cadeaux doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la délégation du bureau en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur, aucune mesure de publicité n'est explicitement explicitement prévue, à la différence des invitations à l'étranger. Le présent amendement tend à combler cette lacune. Il s'agit d'un simple complément au regard de la transparence. Mes chers chers collègues, nous aurons de toute façon une réflexion de fond plus large à mener lors du prochain renouvellement du Sénat, afin de moderniser notre règlement interne pour y introduire plus de transparence et un certain nombre d'innovations démocratiques. Quel

notre assemblée, qui a pris de l'avance dans ce domaine et qui exige depuis longtemps la transparence sur les cadeaux, continuer à assumer sa fonction sans créer une deuxième procédure qui s'ajouterait à la première.

prévoit déjà la transparence pour les invitations d'une valeur supérieure à 150 euros. Les cadeaux doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la délégation du bureau en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur. Il n'y a donc pas de raison de prévoir des mesures de publicité supplémentaires. Le Gouvernement émet

de la liste des documents non communicables aux citoyens les décisions de l'exécutif et de permettre, en particulier, la publicité des délibérations ministérielles et des réunions interministérielles. Cet amendement conservait le principe de non-communicabilité des documents préparatoires, et préservait les garanties protégeant le secret défense, la politique extérieure de la France et la sûreté de l'État.

déclaré irrecevable en commission des lois ce matin, au motif qu'il serait un cavalier législatif au sens de l'article 45 de la Constitution, et donc hors sujet. Je rappelle qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 48 du règlement du Sénat, « les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, en première lecture, s'ils présentent un lien, même indirect, avec le texte en discussion ». Dès lors, nous ne pouvons pas débattre de l'opacité des décisions de l'exécutif en raison de l'opacité des décisions d'irrecevabilité de nos amendements contre lesquelles les parlementaires Déclarer irrecevable un amendement d'initiative parlementaire, c'est empêcher le parlementaire de mener à bien sa mission. C'est inacceptable en général, et plus encore aujourd'hui, compte tenu du sujet qui nous réunit.

Je demande donc qu'à l'avenir l'article 48 de notre règlement sur le droit d'amendement soit respecté à la lettre et qu'il n'en soit plus donné une interprétation restrictive. J'ai bien entendu la réponse du président de la commission des lois à Mme la présidente Assassi. Mais si le Gouvernement oublie

L'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit que « Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication » avec les parlementaires et les organes des assemblées. Il est proposé de renforcer la transparence des documents fournis par les représentants d'intérêts, ainsi que des rencontres et rendez-vous organisés par ces mêmes représentants en demandant au bureau de chaque assemblée de prévoir des mesures de publicité, le principe de cette transparence étant posé par la loi. Il s'agit là d'un point essentiel permettant de lever les suspicions, très fortes actuellement, autour de l'influence réelle des. En effet, si chaque groupe d'intérêts- public, privé, étranger, associatif, ONG -voyait les communications qu'il adresse aux parlementaires, notamment lorsqu'il s'agit de propositions d'amendements prérédigés, rendues publiques, et que l'on puisse dès lors juger de l'adaptation ou de la reprise qui en est faite et des arguments déployés pour les défendre, alors nous pourrions lever tout ou partie du fantasme qui existe autour de ces et prouver à nos concitoyens que nous faisons preuve d'indépendance

ce que fait le bureau du Sénat depuis longtemps et, à cet égard, il a mis en oeuvre des règles pour l'accès des au Sénat. Il lui est loisible de préciser encore ces règles. Nous savons, par ailleurs, que la loi contre la corruption présentée par M. Sapin voilà quelques mois a permis la mise en place d'un registre des représentants d'intérêts. Attendons un peu avant de le réformer.

à ce stade.

les activités de conseil exercées à l'issue d'un mandat parlementaire afin d'éviter tout soupçon. En effet, cette durée correspond à celle de l'indemnité différentielle de fin de mandat à taux plein des parlementaires. Il n'en résulterait donc pas de perte de revenu pour le parlementaire concerné si le conseil était son activité principale avant sa prise de fonctions.

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, a apporté une définition des « représentants d'intérêts ». Aux termes de l'article 25 de cette loi, « sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Idu titre I du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication » avec des responsables politiques. Toutefois, cet article prévoit un certain nombre d'exceptions. Cet amendement tend à les supprimer, sauf dans le cas des élus dans l'exercice de leur mandat, et des partis et groupements politiques dans le cadre de leur mission. Les exceptions que nous souhaitons supprimer sont les suivantes c) les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs d) les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes » ; « e) les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts

parlementaire dans lequel nous devrions faire notre travail en évitant absolument d'être contaminé par tout contact impur avec les représentants de la société civile. À un moment, derrière cette forme de puritanisme, on peut suspecter la fausse dévotion

de parler et d'écouter les représentants de la société civile. Bien sûr ! Nous procédons à de très nombreuses auditions. Les intérêts économiques ont vocation à être entendus, comme les intérêts sociaux. Les organisations syndicales de fonctionnaires, les associations à objet cultuel, les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leur statut, visées par l'amendement de notre collègue Labbé, sont des organisations qui ont été, à dessein, exclues au cours d'un travail parlementaire très approfondi qui date de moins de six mois. Je rappelle que notre assemblée n'a pas changé de composition depuis et s'est exprimée très clairement sur ce sujet. Je ne vois pas pourquoi on remettrait en cause notre propre vote six mois après.

de revenir sur certaines exceptions qui, pour les raisons expliquées par M. le rapporteur, nous semblent pleinement justifiées. C'est la raison pour laquelle, aucune nécessité n'apparaissant immédiatement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Cet amendement vise ainsi à imposer la transparence aux relations entre les représentants d'intérêts et les parlementaires dans le cadre de la confection de la loi.

et c'est donc à regret que je vais émettre un avis défavorable. En effet, je ne voudrais pas que, au fil de ce débat, nous en arrivions à faire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique une sorte de Léviathan devant traiter des questions les plus diverses, ... Très bien ! ... alors que sa vocation est d'enregistrer nos déclarations de patrimoine et d'intérêts ainsi que celles des présidents d'exécutifs locaux, et de s'assurer que, pendant notre mandat, nous ne nous sommes pas enrichis de manière illicite. De grâce, ne mettons pas cette Haute Autorité à toutes les sauces ! Elle a pris le temps de se mettre en place, il a été difficile pour elle de réunir les moyens nécessaires à son activité. Progressivement, elle atteint son régime de croisière. Elle n'a donc pas vocation à servir à tout, même si, je le reconnais, il serait extrêmement intéressant pour chacun d'entre nous, comme pour le public en général, que l'origine des amendements rédigés par les groupes d'intérêts soit tout simplement

qui sont chargés de fixer les règles d'accréditation et d'entrée au sein de leurs chambres respectives. Cet amendement a pour but d'inciter le Sénat et l'Assemblée nationale à prohiber, dans leurs règlements, l'attribution d'un accès permanent à des représentants d'intérêts. En effet, il n'est pas justifiable que des ou des représentants de se promènent dans nos couloirs sans avoir pris rendez-vous avec un parlementaire, dans l'unique but de glaner des informations ou d'exercer des pressions.

présenté d'amendement visant à les interdire, monsieur Labbé, il faut bien qu'ils servent à quelque chose et qu'ils représentent les intérêts légitimes des secteurs économiques ou des professions qu'ils défendent. Au sein de notre assemblée, l'organisation du travail parlementaire relève non de la loi mais du bureau. Nous admettons la présence, en certains lieux, de représentants de groupements d'intérêts, ce qui offre la possibilité de les rencontrer. Ces rencontres sont légitimes, chacun en France a le droit d'approcher le Parlement. Ce qui est interdit, ce sont la corruption, la prévarication, les conflits d'intérêts. Pour ma part, je revendique la possibilité de représenter les intérêts des forces vives et donc de ne pas leur interdire l'accès au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je suis, sur le fond, tout à fait hostile à cet amendement.

Je partage évidemment l'analyse portant sur le caractère législatif de telles propositions, la loi n'a pas à intervenir sur ce terrain.

Il reste peu d'espace au travail parlementaire, mes chers collègues. Il en a de moins en moins ! Ce n'est pas à nous de rogner constamment le champ de la responsabilité propre de chaque assemblée.

Je me sens obligé d'expliquer un peu plus précisément

! Monsieur Bertrand,

on prévoit que, une fois nommée, la personne ne peut délibérer sur les questions intéressant une société

on atteint des résultats non souhaitables. Par exemple, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est nommé en conseil des ministres, conformément à l'article 13 de la Constitution ; or cette disposition interdirait que l'on choisisse quelqu'un qui a dirigé une filiale

À quand une pause législative ? Je crois que nous aurions mieux fait de la faire sur ce sujet et de prendre le temps de la réflexion avant de légiférer comme nous le faisons en ce moment. Très

les intérêts politiques les plus importants et la très haute administration. C'est cela, la France ; c'est cela, le système ! J'ai d'ailleurs essayé d'en dire quelques mots dans la discussion générale. Et

aux électeurs, tout véritable pouvoir. C'est là qu'est l'origine profonde de cette opposition, ce fossé qui est en train de se creuser entre nous et nos électeurs.

recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts. Le Gouvernement y voit deux obstacles majeurs. En premier lieu, il nous semble que ces dispositions ne peuvent figurer dans la loi sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs,

à la transparence de la vie publique a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer non seulement les modalités de son application, mais aussi « les conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement En précisant que le registre doit mentionner les cas dans lesquels un membre du Gouvernement s'abstient de participer à la délibération du conseil des ministres, l'article 2 nous contraire à la Constitution, parce qu'il intervient dans une matière qui est au coeur de l'organisation du pouvoir exécutif et qui relève donc, par principe, de la seule compétence du pouvoir exécutif,

le texte de la commission est très large et pourrait précisément entrer en contradiction avec le principe selon lequel ne sont pas communicables les « documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement Enfin, et en tout état de cause, les membres du Gouvernement connaissent déjà des mécanismes de prévention des conflits d'intérêts. À cet égard, la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique indique, dans son article 1, que les membres du Gouvernement « exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts

a été précisément pris en application de l'article 2 de la loi précitée. Aux termes de ce décret, lorsque le Premier ministre se trouve en situation de conflit d'intérêts pour l'exercice de certains de ses pouvoirs, il délègue ceux-ci au ministre premièrement nommé dans le décret relatif à la composition du Gouvernement. Lorsque c'est un ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, il en informe le Premier ministre. Un décret détermine ensuite les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé. Un mécanisme similaire existe enfin lorsqu'il s'agit d'un membre du cabinet qui est placé auprès d'un ministre. Ce système est tout à fait est tout à fait respectueux du principe de la séparation des pouvoirs. Il paraît suffisant et effectif. À titre d'illustration, comme vous le savez, le décret du 29 mai 2017, qui a été pris en application de l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959, en est un exemple. Par celui-ci, la ministre des solidarités et de la santé, Mme Agnès

la commission ? La commission s'en tient à son texte. Il est tout de même singulier que le Gouvernement, qui a beaucoup de bonnes idées pour assurer la transparence du travail parlementaire, soit aussi frileux quand il s'agit, symétriquement, d'améliorer celle du travail gouvernemental.

pourrait accueillir avec davantage d'ouverture d'esprit un tel amendement. D'ailleurs, de manière générale, nous nous sommes efforcés de tenir la balance égale entre l'exécutif et le législatif. C'est tout à fait normal ! Vous utilisez quelques arguments de droit. Vous

ce que n'est pas le conseil des ministres, qui est un organe constitutionnel tout à fait différent. Telle est la raison pour laquelle je maintiens la demande de suppression Ayant siégé dans un conseil municipal comme au conseil des ministres, j'oserai, comme vous, madame la garde des sceaux, me prévaloir d'une certaine expérience dans ce domaine. Si les assemblées municipales et le conseil des ministres ne sont pas de même nature, ce n'est pas une raison suffisante pour écarter l'application de règles communes quand il s'agit de conflits d'intérêts. Tout à fait ! Madame la garde vous rappeler que la loi de 2013 fait injonction à l'exécutif de faire cesser les conflits d'intérêts et que le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à y redire. Dans ces conditions, je n'imagine pas qu'il puisse s'opposer à une mesure améliorant la transparence du fonctionnement du conseil des ministres

qui nous empêcherait de légiférer sur toute matière qui relève de l'exercice du pouvoir exécutif. Cela nous conduirait à des absurdités. Je crois donc vraiment que la commission des lois a bien fait de suivre son rapporteur.

vous me pardonnerez de faire à nouveau référence au Conseil constitutionnel, qui, dans une décision de 2011, a clairement précisé qu'il

La séance est suspendue.